j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Yves Goussebaire-Dupin, qui fut sénateur des Landes de 1983 à 1992. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

territoriales (CGCT), il vise à supprimer l'obligation de pose de la première plaque de numéro à la charge de la commune, afin d'alléger le coût et le temps de mise en oeuvre par les communes d'un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales. Le besoin de pose des plaques de numéro et de voies est laissé à l'appréciation des communes, qui sont les plus à même de juger de leur nécessité. Cet amendement tend également à prévoir que les communes garantissent l'accès aux informations concernant les adresses au format standard en vigueur, le format de la base adresse locale (BAL), en alimentant le point d'accès national mis en oeuvre dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, c'est-à-dire la base adresse nationale (BAN), afin notamment de faciliter le déploiement et la commercialisation du très haut débit sur l'ensemble du territoire, mais aussi pour des raisons de sécurité. Les conditions Les conditions de mise en oeuvre, en particulier du point de vue du délai, des obligations d'adressage et de remontée d'information sur les adresses seront définies par un décret en Conseil d'État.

les conseils municipaux ont compétence pour numéroter les immeubles et dénommer les rues ; c'est une compétence obligatoire pour les communes de plus de 2 000 habitants, qui constituent ainsi une base d'adresses.

l'intermédiaire des maires, doivent communiquer à de nombreuses administrations- fiscales, environnementales ou d'infrastructure -les mêmes données, dans des formats différents.

Si la démocratie locale doit naturellement, à titre principal, s'exercer avec des élus présents dans les hémicycles, il serait regrettable de se priver, hors période de crise, de la faculté d'organiser ponctuellement, au regard de considérations locales, des réunions à distance. Ainsi le

L'usage de la téléconférence est strictement encadré, afin de garantir le bon déroulement des réunions et le respect des règles qui s'imposent déjà aux réunions des organes délibérants des collectivités.

Ces dispositions permettent la réunion de l'organe délibérant soit en plusieurs lieux distincts, soit par visioconférence, en y ajoutant néanmoins une limite : le conseil doit se réunir en présence au moins une fois par semestre. En outre, la réunion doit se tenir en présence notamment pour l'élection du président et le vote du budget primitif. Les mesures proposées prévoient que les conditions de publicité doivent offrir au public les mêmes facilités d'accès qu'aux conseillers. Ainsi, une réunion, qu'elle soit partiellement ou intégralement tenue par visioconférence, doit faire l'objet d'une retransmission en direct sur le site de la collectivité ou de l'EPCI. En cas de réunions tenues depuis plusieurs sites distants, tous ces sites doivent être ouverts au public. Les modalités d'organisation des réunions sont précisées sur la convocation

de la loi. Or ces structures publiques peuvent couvrir des territoires géographiques importants et souhaitent pouvoir utiliser la visioconférence, outil de dématérialisation et de développement durable. Quel est l'avis de la commission ? Ces amendements

et qui ont démontré leur intérêt et leur utilité pour éviter de trop nombreux déplacements et permettre au plus grand nombre d'élus de participer. Cette possibilité avait été ouverte pour les seuls EPCI à fiscalité propre

en particulier pour les décisions les plus importantes- je pense au vote du budget -, et prévoir que l'assemblée délibérante se réunisse physiquement au moins une fois par semestre.

Cette modalité a été testée avec succès lors du premier confinement dans de nombreuses collectivités. Sa prolongation permettrait de faciliter l'accès des administrés aux décisions de nos collectivités.

l'entrée en vigueur et la conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Une large consultation a été menée avec les associations d'élus, notamment l'Association des maires Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et le Conseil d'État seront saisis du sujet d'ici à la fin du mois. En l'état du droit, la publicité des actes communaux doit être assurée sur papier leur publicité sous forme électronique n'est possible qu'à titre facultatif et complémentaire. Il sera donc proposé de renforcer le recours à la dématérialisation de la publicité des actes des communes, tout en tenant compte des moyens des plus petites communes. Ainsi, les régions, les départements et les communes de 3 500 habitants et plus devront assurer la publicité de leurs actes sous forme électronique uniquement ; d'ailleurs, la plupart le font déjà. Les communes de moins de 3 500 habitants se verront offrir le choix entre trois options la publicité par voie d'affichage, la publicité par voie de publication sur papier et la publicité par voie électronique. Elles devront opter pour l'une de ces solutions afin de sécuriser, pour tous, l'entrée en vigueur des actes locaux

Cet amendement a pour objet de sécuriser les moyens des groupes politiques des collectivités territoriales. En réponse aux questions soulevées à l'occasion de l'installation des nouveaux conseils régionaux et conseils départementaux ou lors de contrôles de chambres régionales des comptes,

afin de permettre l'exercice de la mission de tous les élus dans le respect du pluralisme d'expression au sein de l'organe délibérant, le maire ou le président peut au sein de ces collectivités, dans les conditions fixées par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe d'élus, affecter à ces groupes une ou plusieurs personnes. L'organe délibérant ouvre alors, par délibération au budget de la collectivité, les crédits nécessaires à ces dépenses, dans la limite d'un plafond dans la limite d'un plafond fixé à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux élus de l'organe délibérant- Toutefois, le texte actuel relatif à ce dispositif institutionnel ne précise pas si ce montant doit être compris comme intégrant les charges sociales auxquelles sont soumises ces indemnités

ont fait l'objet de remarques de la Cour des comptes. L'objet de cet amendement est donc de préciser cette disposition et de sécuriser juridiquement les décisions des collectivités concernées, en indiquant que le montant doit s'entendre étant égal à 30 % des indemnités, charges comprises. Cette mesure rassurera les collectivités territoriales qui sont en train de délibérer et d'aménager le fonctionnement de leur organe

en sus des communes et des groupements de communes, et permet à l'ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. S'agissant de déléguer un droit de préemption sur tout ou partie d'une aire d'alimentation de captages et non pas seulement lors d'opérations ponctuelles d'aliénation, il semble préférable d'en réserver l'exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents, qui doivent en conserver la pleine maîtrise. Les titulaires précités, qui demeurent les garants de l'intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le foncier acquis, le cas échéant, à des régies, si cette rétrocession se révèle nécessaire. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l'article L. 2221-10 du CGCT. La parole est à M.

peut tout à fait déléguer l'activité de gestion du captage. Toutefois, la prise en charge de l'acquisition des sols, avec les aspects stratégiques que cela comporte, doit, selon nous, rester de la seule responsabilité des collectivités territoriales ou de leur groupement.

destinées à la consommation humaine- il s'agit de l'article L. 218-1 et suivants du code de l'urbanisme -, en considérant l'avis du Conseil d'État pour les rendre applicables. La délimitation de ce droit de préemption, effectuée par l'autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires, portera sur des surfaces agricoles dans l'aire d'alimentation de captages utilisée pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, sur tout ou partie de ces territoires. Les aires d'alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont souvent de grande qualité agronomique pour la production agricole.

tout en appréhendant au mieux l'activité agricole, son évolution nécessaire, et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires. Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu'il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les Safer, suffisamment en amont dans le cadre des projets locaux. Il s'agit d'articuler les objectifs poursuivis le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au premier alinéa du I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Les objectifs cités sont la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture par l'installation et la consolidation d'exploitations agricoles. Cet amendement tend à s'inscrire dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers,

Pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, il est indispensable que les acteurs fonciers des territoires travaillent de concert, tout particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les Safer.

et 1637 rectifié visent à supprimer la faculté de déléguer l'exercice du droit de préemption à un établissement public local. Il arrive fréquemment qu'une commune, un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat délègue tout ou partie de sa compétence en matière d'eau potable à un établissement public créé à cet effet. Dans ce cas, la compétence n'est pas exercée en régie directe, mais par l'intermédiaire d'une régie personnalisée. L'article 60 du projet de loi prévoit que, dans ce cas, l'autorité compétente puisse aussi déléguer à cet établissement public l'exercice de son droit de préemption

à soutenir les libertés locales, imposer aux communes ou à leurs groupements de conventionner avec la Safer pour exercer le droit de préemption de terrains agricoles. S'il faut que les collectivités discutent, y compris avec la Safer,

présenter l'amendement n° 171 rectifié Si la protection de la ressource en eau doit, dans certains secteurs, s'accompagner de changements de pratiques agricoles des clauses environnementales proposées au preneur en place, il est essentiel que la nature de ces clauses et leur objet puissent être appréhendés au regard des impacts qu'elles engendrent sur l'exploitation agricole de l'occupant des parcelles concernées. Un accompagnement par une chambre d'agriculture susceptible d'apporter des conseils pédologiques, technico-économiques technico-économiques et agronomiques serait de nature à garantir les résultats attendus en matière de qualité de l'eau, tout en préservant un équilibre économique pour le locataire en place.

puissent rétrocéder sans délai les parcelles acquises. Il convient donc d'imposer un délai de conservation dont la durée équivaut à celui de la durée minimale d'un bail rural.

L'amendement vise à introduire une précaution juridique en relation avec leur objet d'intérêt public, en prévoyant que les propriétés restent dans le patrimoine de la collectivité ou de l'établissement qui les a acquises pendant au moins la durée d'un bail agricole.

au-delà des contraintes imposées dans les dispositions régissant l'acte de vente, le propriétaire dispose du bien qu'il a acquis. Or ces amendements prévoient qu'un EPCI ou une commune qui aurait

me semble assez compliquée puisqu'une commune ou un EPCI n'a pas vocation à exploiter directement des terres agricoles. On ne peut pas imposer à une collectivité de laisser des terrains en friche pendant neuf ans au prétexte qu'elle ne peut pas les confier

d'une acquisition contrainte avec un objectif d'intérêt public. Aussi, logiquement, la collectivité ne s'est pas trompée en achetant ce terrain par voie de contrainte : c'est pour elle une nécessité. madame la rapporteure, mais l'amendement ne tend aucunement à empêcher la collectivité de donner à bail ce bien et de le rendre inutile sur le plan agricole. C'est bien le transfert de propriété qui est problématique. Il me semble que la prudence constitutionnelle consisterait plutôt à ne pas trop se risquer sur ce sujet.

Elles se traduisent par l'inscription dans un contrat d'obligations ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Ce régime est donc totalement en phase avec l'esprit des objectifs environnementaux et climatiques que la France se fixe. Or les rapporteurs ont supprimé ce régime, au motif qu'il était « extrêmement lacunaire

Dans un rapport du Gouvernement rendu au Parlement en janvier 2021 sur ces obligations, aucune remise en cause de ce dispositif n'a été mise en avant. Si le Gouvernement y reconnaissait que « l'absence de mécanisme de suivi de la signature de ces contrats rend difficile l'existence d'une vision nationale de la mise en oeuvre » de ces obligations, il n'en remettait nullement en cause l'existence et la pertinence. Il précisait même, en conclusion, que si des évolutions du mécanisme des obligations peuvent être envisageables, telle décision « semble en tout état de cause prématurée compte tenu du manque de recul sur l'utilisation de cet outil dont elle serait de nature à changer la philosophie ». Nous proposons tout simplement de ne pas supprimer ce régime. La parole est à M. Joël Labbé,

coécrit par Frédérique Tuffnell, députée de Charente-Maritime, et notre excellent ancien collègue Jérôme Bignon, qui était un véritable défenseur des zones humides et de la qualité de l'eau. Ce rapport préconisait de développer des exonérations fiscales appropriées pour le développement des obligations réelles environnementales afin de préserver les zones humides. J'évoquerai aussi l'avis du Comité national de la biodiversité sur la « Stratégie nationale pour les aires protégées 2030 », ou encore une récente note de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, laquelle plébiscite également

environnementales a été introduit par la loi Biodiversité. Il est au coeur du désormais fameux article 2 de la Charte de l'environnement, lequel dispose que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous nous opposons à ce que toute personne publique ou privée puisse apporter un concours financier aux ouvrages et aménagements de contrat de concessions autoroutières. En effet, puisque ces contrats existent, les concessionnaires doivent se rémunérer sur les péages et ne pas attendre des subsides des collectivités de l'État ou des opérateurs privés. Actuellement, les conditions de concessions sont telles que la rentabilité pour les actionnaires justifie de refuser tout concours public ou privé au financement des ouvrages. Pour autant, nous restons sur une position de principe : nous souhaitons que l'État stratège prenne enfin ses responsabilités, et engage une renationalisation des concessions autoroutières et la création d'un établissement public « Autoroutes de France 100 % public, afin de garantir le respect du patrimoine payé par l'argent des contribuables publics et pour l'intérêt général. Le présent article permet à des personnes privées de concourir au financement des aménagements dans le cadre des concessions autoroutières. Ainsi, vous permettez à une société comme Disney de financer, demain, des autoroutes pour rejoindre son parc d'attractions, à Marne-la-Vallée. Je pourrais prendre d'autres exemples ... Ce mélange des genres entre intérêt public et intérêts privés ne nous semble pas souhaitable. Il crée une confusion préjudiciable à l'action publique et encourage une forme de privatisation de l'aménagement, qui ne répondrait pas aux besoins exprimés par la population, mais aux intérêts économiques et financiers du territoire. Nous nous opposons à de telles pratiques et souhaitons, à l'inverse, remettre de l'intérêt général et de la morale dans la gestion des infrastructures nationales, notamment autoroutières. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement

utiles au développement économique local, tout en évitant une hausse des péages. L'intention initiale n'était pas d'interdire le financement d'ouvrages ou d'aménagements des réseaux concédés par des tiers, mais plutôt d'encadrer

Nous avons certes des marges de progrès en termes de contrôle et de régulation des concessions autoroutières, mais je ne suis pas favorable à interdire le recours à cet outil pour le financement de nouvelles infrastructures. L'avis est donc défavorable.

si l'abattage d'un ou plusieurs arbres est interdit, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres représente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres. Toutefois, sur ce fondement, des difficultés locales apparaissent des difficultés locales apparaissent qui conduisent à des incertitudes et à des contentieux entre conseils municipaux et autorités préfectorales. Si le présent article clarifie lesdits régimes en désignant le préfet de département comme autorité administrative compétente, convaincu de la pertinence du couple maire-préfet, qu'il faut respecter les prérogatives des communes et renforcer le dialogue. Dans la mesure où nos communes représentent l'échelon le mieux à même d'estimer la dangerosité de certains arbres et de décider de leur abattage, le représentant de l'État

: La parole est à M. Jacques Fernique. « Je considère que les alignements d'arbres le long des voies de communication offrent un paysage de qualité, en même temps qu'ils protègent les infrastructures, en particulier en stabilisant leurs bas-côtés. Je suis donc évidemment favorable, par principe,

350-3 du code de l'environnement, aujourd'hui dans le collimateur de cet article 62. Je veux bien sûr parler de l'actuelle ministre de la transition écologique, Barbara Pompili. Notre amendement tend à la suppression de l'article 62, pour en rester au droit en vigueur. Le maintien de l'article L. 350-3 apparaît essentiel sur bien des aspects. La facilitation de l'abattage des allées et alignements d'arbres qui bordent nos voies de communication pour favoriser la réalisation d'infrastructures relève d'une logique d'aménagement à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, de préservation du patrimoine et de la nécessité de préserver ces arbres si importants contre le réchauffement, comme le récent paquet climat européen vient de le réaffirmer fortement.

eux, n'ont, semble-t-il, d'autres défenseurs que moi-même et il apparaît que cela ne compte pas. La France n'est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture, et, quelle que soit l'importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. » Après celle de Barbara Pompili, je soumets cette citation de George

d'abattage d'un arbre situé dans une allée d'arbres. Il permet ainsi de mettre fin à des situations dans lesquelles les communes se trouvaient à la fois juge et partie, puisqu'elles étaient amenées à autoriser des atteintes aux allées d'arbres pour permettre la réalisation de travaux routiers dont elles étaient maîtres d'ouvrage. La rédaction adoptée en commission conserve le régime de protection prévu par l'article 62 en précisant qu'il s'applique aux voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des voies privées, afin de garantir le respect du droit de propriété. ailleurs, l'inclusion des voies privées dans le dispositif pourrait engendrer des effets pervers : comme l'a reconnu la jurisprudence administrative, les propriétaires peuvent décider à tout moment d'interdire l'ouverture au public de voies qu'ils possèdent. soumettre les allées d'arbres bordant des voies privées à ce régime peut donc conduire les propriétaires à fermer ces voies à l'accès du public, ce qui n'est pas souhaitable. Enfin, en ce qui concerne les mesures compensatoires, l'article 62 prévoit qu'elles

ne vise ainsi plus les allées d'arbres et alignements d'arbres qui « bordent les voies de communication », mais ceux qui bordent les voies « ouvertes à la circulation publique ». Les auteurs de cet amendement sont assez dubitatifs sur la portée de cette modification. Ils s'inquiètent qu'elle ne revienne à restreindre les zones de protection des allées et alignements d'arbres. En conséquence, ils proposent une nouvelle rédaction, plus large, afin de s'assurer que le champ d'application ne soit pas

ou le passage destructeur d'engins de travaux. Ne plus protéger les voies privées revient concrètement à ne plus protéger toute voie non ouverte à la circulation publique : chemins de halage, voies sur berges des canaux et rivières, chemins ruraux ... Autant de lieux où ces arbres ont toute leur place et jouent un rôle d'autant plus important qu'ils font déjà partie d'un ensemble naturel. Cela déstabiliserait encore davantage les écosystèmes alentour. Notre amendement, simple et cohérent, concerne les types de voies qui devraient faire partie du périmètre de protection, à savoir les voies ouvertes ou non à la circulation publique, les chemins publics ou privés, les canaux et voies d'eau, les voies ferroviaires. Il tend à énumérer de façon plus exhaustive les voies sur lesquelles les arbres font l'objet d'une protection spécifique.

il revient sur la rédaction adoptée en commission, qui exclut spécifiquement les voies privées de ce dispositif afin de garantir le respect du droit de propriété. En revanche, le II dudit amendement permet de clarifier la rédaction du premier alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.

L'encadrement des mesures compensatoires prévues perd en précision : il ne comprend plus un volet en nature- plantations -et un volet financier destinés à assurer l'entretien ultérieur de la zone d'arbres, comme le prévoit la législation actuelle. disposition est complexe, mais elle est nécessaire. Le préfet statuera simplement sur « le caractère suffisant » des mesures de compensation qui devront accompagner la demande d'autorisation. Introduire de multiples dérogations pour l'abattage des allées d'arbres en cas de travaux, et laisser le préfet décider du sort des arbres face à des projets d'aménagement, interroge. Je mets en garde contre les risques et conséquences graves que cela implique.

? Établir l'impossibilité technique pour le pétitionnaire de conduire des travaux sans porter atteinte aux allées d'arbres me semble difficile à mettre en oeuvre pour les communes et risque de conduire à de nombreux blocages pour les projets d'infrastructures. de l'amendement n° 1273 comprend des ambiguïtés puisqu'elle prévoit la démonstration d'une impossibilité technique à agir sans porter atteinte à l'arbre pour toutes les demandes d'autorisation. Or il conviendrait d'exclure les cas où l'arbre présente un danger pour les personnes ou un danger sanitaire pour les autres arbres. Enfin, en ce qui concerne les compensations, cet amendement me semble déjà en partie satisfait puisque l'article 62 prévoit la présentation des mesures compensatoires dans le cadre de la demande d'autorisation.

d'arbres. Lorsque l'état sanitaire de l'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou encore un danger pour les autres arbres, le Gouvernement propose de recourir à une procédure de simple « déclaration préalable » auprès du préfet de département plutôt qu'à une procédure d'autorisation, laquelle nécessite plusieurs mois d'instruction. permettra d'alléger les procédures à mettre en oeuvre pour les communes et les services de l'État et de raccourcir les délais d'intervention. En revanche, lorsque la demande a pour origine un projet d'aménagement, le Gouvernement propose de conserver la procédure d'autorisation formelle auprès du préfet de département. Cela me semble judicieux, car il importe, dans ce cas de figure, que le préfet puisse apprécier la nécessité des mesures envisagées. Cette proposition me semble aller dans le sens d'une simplification des procédures pour les collectivités, tout en conservant des exigences de contrôle des atteintes portées aux alignements d'arbres

En vertu dudit article L. 350-3, le préfet doit pouvoir apprécier la réalité de ce danger, qui doit être démontrée par la commune. En supprimant le contrôle du préfet, rien ne permet d'assurer le respect des conditions dérogatoires pouvant conduire à l'abattement d'un arbre. De plus, il me semble que nous retrouverions alors la situation de conflit d'intérêts qui a donné lieu à des contentieux au niveau local et qui a justifié l'intervention du législateur visant à préciser l'autorité compétente

haies et alignements constituent des éléments non négligeables des continuités écologiques et contribuent à la qualité de l'air, aux fonctionnalités écologiques des sols, au stockage du carbone et à la qualité paysagère. également une biodiversité importante, source de résilience pour nos territoires. Au même titre que les agriculteurs, les collectivités ont un rôle important à jouer pour la bonne fonctionnalité de ces linéaires de haies et d'alignements d'arbres en bord de voirie dont elles entretiennent la partie qui jouxte la route. Aujourd'hui, si de bonnes pratiques de gestion de ces linéaires existent, elles sont encore trop peu développées, car trop souvent méconnues des collectivités. Pourtant, ces bonnes pratiques sont recensées et ne constituent pas une contrainte pour les élus locaux. Elles peuvent d'ailleurs

de bois énergie. À titre d'exemple, des conseils départementaux mettent en place des programmes de valorisation d'une ressource bois énergie locale, notamment leur gestion durable des haies en bordure de voirie. Il ne s'agit donc pas ici de contraindre les collectivités, mais de leur envoyer un signal fort sur l'intérêt de la gestion de ces espaces. Nous proposons un délai de deux ans et demi pour laisser aux collectivités le temps de s'adapter. est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ? Je ne suis pas favorable à l'instauration d'une telle obligation pour les communes, car elle ne va pas dans le sens de la simplification. Les communes sont libres de mettre en place des outils de gestion durable des allées d'arbres ou de haies, si elles le souhaitent

c'est que chaque année la France perd plus de 11 000 kilomètres linéaires de haies, et ce malgré des opérations de plantations- c'est un résultat net. De bonnes pratiques en matière d'urbanisme associées à la création d'un dialogue au niveau local permettent pourtant de préserver efficacement le linéaire de haies et d'alignements d'arbres existant, et même de le développer. Ces bonnes pratiques sont déjà mises en oeuvre par de nombreuses collectivités. Afin d'encourager davantage les élus locaux à se saisir de ces bonnes pratiques et à reconnaître le rôle majeur de la haie et des alignements d'arbres comme outils de transition écologique, nous proposons de mentionner explicitement les haies, alignements d'arbres et trames bocagères dans le code de l'urbanisme, tant à l'échelle des principes généraux dudit code

aux élus, aux agriculteurs et à l'ensemble de nos concitoyens dans le sens de la construction d'un dialogue local. L'adoption de cet amendement ne changerait pas le droit existant et ne créerait pas de contrainte pour les élus locaux.

à propos de l'amendement précédent, il me semble qu'imposer dans la loi de nouvelles obligations aux communes sur ce sujet n'est pas souhaitable. Les élus locaux n'ont pas besoin du législateur pour mettre en place les outils nécessaires à la préservation de ce patrimoine paysager ni pour engager le dialogue avec d'autres acteurs locaux concernés comme le public ou les agriculteurs. Par ailleurs, Par ailleurs, il me semble que cette proposition est en réalité satisfaite par le code de l'urbanisme. L'article L. 101-2 dudit code impose déjà aux collectivités un objectif de protection des sites, des milieux et des paysages naturels dans leurs politiques d'urbanisme. L'article L. 141-4 permet la prise en compte, dans l'élaboration du document d'orientation et d'objectifs du PLU, de la préservation et de la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'article L. 151-19 permet quant à lui d'intégrer au règlement du PLU la conservation des éléments du paysage. L'article L. L'article L. 151-23 permet d'identifier, dans ce même règlement, les éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique.

loi. Actuellement, la protection des milieux naturels, de la biodiversité, des écosystèmes, ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques font déjà partie des principes édictés par le code de l'urbanisme des SCoT. Le code de l'urbanisme prévoit également plusieurs outils permettant de protéger le patrimoine arboricole, les haies et les trames bocagères dans le cadre des PLU, pour des raisons écologiques, architecturales et patrimoniales. De d'autres dispositions permettent d'imposer des plantations et des emplacements réservés pour des trames vertes ou encore le classement de secteurs au titre des espaces boisés classés,

et l'égalité d'accès au service de distribution de gaz, à faciliter et à accélérer le transfert des conduites d'immeubles et conduites montantes au réseau public de distribution de gaz, en permettant

De surcroît, l'application pratique des dispositions de la loi précitée afférentes aux colonnes montantes électriques a révélé que le lissage des transferts des colonnes sur une période suffisamment longue permettait d'éviter un transfert massif au lendemain de l'échéance et de recueillir avant le terme les retours d'expérience, de manière à pouvoir adapter la procédure si nécessaire.

sans détruire ». Afin de rééquilibrer le partage des responsabilités, Michel Canévet et les cosignataires de cet amendement proposent de préciser que l'exécutant des travaux ou le responsable de projet sont tenus de respecter l'ensemble de la réglementation anti-endommagement pour ne pas se voir imputer la responsabilité d'un dommage sur un ouvrage.

Quant à l'amendement n° 978 rectifié, qui vise à modifier les conditions d'engagement de la responsabilité dans le cas d'endommagements accidentels, les évolutions suggérées sont de nature essentiellement réglementaire, puisqu'il serait fait mention de la réglementation anti-endommagement avec des références très précises aux prescriptions et recommandations techniques ainsi qu'aux affleurants ou aux grillages. En outre, ces évolutions introduiraient de la complexité, ce qui ne serait pas nécessairement favorable aux gestionnaires de réseaux, dont la responsabilité a- il est vrai -été rééquilibrée par le présent article au profit des entreprises. Je vous demande donc, mes chers

de comptage de gaz au réseau public de distribution. À cette fin, le code de l'énergie disposerait que les propriétaires ou syndicats des copropriétaires doivent permettre aux opérateurs des distributeurs de gaz et d'électricité d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz et d'électricité. Or la rédaction actuelle du dispositif est insuffisante pour s'assurer du bon déroulement de ces visites prévues par la loi. En effet, l'accès aux ouvrages de distribution ne saurait être seulement permis : il doit être garanti. Cet amendement déposé par Hervé Marseille a pour objet de modifier la rédaction de l'article L. 126-15 du code de la construction et de l'habitation afin de garantir un accès effectif aux ouvrages de distribution. Dans la mesure où le projet de loi impose la réalisation de visites de bon fonctionnement, il est nécessaire que les syndics garantissent cet accès afin que les gestionnaires de réseaux satisfassent à ces nouvelles obligations. La parole

abonnés de réseaux de chaleur, qui sont eux-mêmes soutenus financièrement par l'État. Cette situation est par ailleurs en totale contradiction avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d'énergie fossile et de développement de la chaleur renouvelable.

en concertation avec les représentants des autorités organisatrices de la distribution d'énergie, de sorte qu'un dialogue territorial permet déjà d'identifier les territoires les plus propices à cet effort de développement. Par ailleurs, l'interdiction de toute concurrence entre les réseaux de gaz et les réseaux de chaleur, d'une part, serait contraire au principe constitutionnel de libre concurrence et, d'autre part, ne dirait rien des autres sources d'énergie. Enfin, sur le plan pratique,

n° 358 rectifié . Cet amendement vise à combler une lacune de l'article du code de l'énergie définissant les communautés d'énergie renouvelable.

disposition proposée contrevient à la définition des communautés d'énergie renouvelable, directement issue de la transposition de l'article 22 de la directive du 11 décembre 2018 sur les énergies renouvelables. elle induirait une différence de traitement entre les communautés d'énergie renouvelable, auxquelles elle s'appliquerait, et les communautés énergétiques citoyennes, qui seraient laissées de côté.

en leur confiant la réalisation du comptage de la production de biogaz dans les zones non desservies par un réseau de gaz naturel. L'ajout de cette nouvelle mission est essentiel pour permettre la mise en oeuvre du dispositif de complément de rémunération pour le biométhane non injecté, destiné à favoriser le développement de la méthanisation sur l'ensemble des territoires. Outre cette précision essentielle relative à la mission de comptage de la production de biogaz,

des contrats d'achat et de complément de rémunération de biométhane, ainsi que de préciser les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect de la réglementation. Si ces dispositions sont accueillies positivement par les gestionnaires de réseaux, elles suscitent l'inquiétude des professionnels du biogaz. Or la période actuelle

dans la mesure où cette enveloppe est normée. Ensuite, elle reviendrait à allouer des moyens importants aux syndicats d'énergie alors que les compétences, elles, seraient toujours largement détenues par les communes ou par leurs groupements, ce qui serait incohérent et, pire, dangereux pour l'investissement local. Il vaut mieux laisser aux communes et aux intercommunalités la faculté de définir, elles-mêmes et librement, les moyens qu'elles entendent conférer aux syndicats d'énergie pour l'exercice de leurs missions. Je demande donc le

d'urbanisme, sans avoir fait l'objet d'aucune consultation préalable des élus locaux. Enfin, cette évolution serait inédite dans notre droit puisque c'est bien la notion de « prise en compte » et non de « compatibilité » qui prévaut en matière de planification, à l'égard des

est encore équipé de lampes à vapeur de mercure, pourtant interdites depuis 2015. En outre, avec 10 millions de points lumineux en France et une consommation énergétique d'environ 5 térawattheure par an, soit 1 % de la consommation électrique nationale, la part de l'éclairage public dans l'empreinte écologique de notre pays est loin d'être négligeable. Le remplacement des matériels faisant appel à des technologies anciennes aujourd'hui obsolètes permet aux collectivités de réaliser d'importantes et rapides économies sur leurs factures d'énergie, et de réduire substantiellement les coûts de maintenance et d'entretien si des automatismes intelligents d'allumage et d'extinction sont associés au remplacement des luminaires. Pour accélérer le renouvellement des réseaux d'éclairage public par des équipements plus performants, il convient de ne pas limiter aux seuls EPCI compétents en matière d'éclairage public l'obligation de prévoir, dans le programme d'actions défini dans le PCAET qu'ils sont tenus d'adopter, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation d'énergie de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.

à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre membres, l'élaboration du PCAET ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique, notamment celle des réseaux d'éclairage public lorsque cette compétence leur a été transférée.

article 7 a bien acté que l'on ne subordonnait plus le programme de maîtrise de la consommation d'énergie de l'éclairage public à la détention de la compétence éclairage public par un EPCI.

Le maire n'est pas forcément informé de cette procédure, alors même qu'il est le garant de l'urbanisation de sa commune et le premier concerné par une évolution à venir sur les exploitations de sa commune. Afin de renforcer l'efficacité de la mise en relation entre cédants et repreneurs, le présent amendement vise à informer systématiquement le maire de la commune lorsqu'un exploitant prévoit d'arrêter son activité dans les trois ans à venir.

de ces déclarations de cessation d'activité. En outre, comme le prévoit le droit en vigueur, l'autorité administrative peut mettre à la disposition du public cette information, et la chambre départementale tient à jour un répertoire départ-installation recensant les exploitations disponibles ou susceptibles de l'être sous trois ans. Dès lors, il ne me semble pas utile d'alourdir la procédure à la charge de l'exploitant dans la loi. Une transmission par la chambre départementale au maire, au même titre qu'à la préfecture,

Cet amendement, déposé par notre collègue Stéphane Demilly, vise à s'assurer que la mission de service public assurée par les chambres d'agriculture se réalise au profit de l'État mais également des régions. régions. Le code rural a confié aux chambres d'agriculture une mission de service public en matière d'installation de jeunes agriculteurs. Or les arbitrages rendus dans le cadre de la prochaine programmation 2023-2027 du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ont pour effet de déléguer aux régions la gestion de la politique de l'installation. Pour s'adapter à ce nouveau contexte et afin que cette mission de service public réalisée par les chambres d'agriculture

à l'Assemblée nationale et sera voté dans les mêmes termes, dans un délai raisonnable. À défaut, il faudra trouver un autre dispositif pour le Haras national du Pin, car nous avons vraiment besoin du transfert. Pour une fois que le département est d'accord avec la région sur un projet

de conformité au raccordement du réseau de collecte des eaux usées dès lors qu'il s'agit d'assainissement collectif. Cette obligation sera faite au moment de la vente de biens immobiliers, comme cela se pratique déjà dans beaucoup de collectivités : il y va de de la qualité de l'eau. Ce dispositif a été mis en place dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 pour reconquérir la qualité de l'eau dans la Seine. l'eau dans la Seine. Vous souhaitez rallonger le délai dont dispose la collectivité pour effectuer ce contrôle. Le délai était d'un mois, vous voulez le faire passer à deux mois.

Le maintien de ce délai permet de ne pas bloquer le marché immobilier et la vente de biens, qui est un exercice compliqué parfois.

serait astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public si son immeuble avait été raccordé.

éventuellement assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 100 euros par jour, le total des sommes résultant de l'astreinte ne pouvant excéder 5 000 euros.

propose de remplacer le dispositif actuel en cas de manquement par le propriétaire à ses obligations au titre du code de la santé publique en matière d'assainissement collectif ou non collectif par un dispositif de mise en demeure avec astreinte. Vous soulignez, madame la rapporteure, que le dispositif actuel serait une sanction déguisée en redevance pour service rendu.

est à M. Claude Kern. Cet amendement tend à décliner la planification régionale au niveau intercommunal sur le modèle de la planification énergétique, afin de permettre une adaptation précise et locale selon les caractéristiques territoriales et les spécificités de l'organisation opérationnelle de la gestion des déchets, en particulier non ménagers.

donner aux EPCI une compétence de planification pour la gestion de l'ensemble des déchets, y compris ceux produits par les industries ou les travaux publics, ne me semble ni simple ni réaliste. Il n'est, à mon avis, pas non plus souhaitable d'imposer un plan local de gestion des déchets aux installations portées par des entreprises.

Un groupe de travail constitué sur le sujet a rendu un rapport en novembre 2018 : le Gouvernement a eu toute latitude pour travailler à l'élaboration d'un projet de loi, ce qu'il n'a pas fait. Le recours à une ordonnance la dernière année du quinquennat nous paraît, dès lors, tout à fait inopportun.

Aujourd'hui, les services de la publicité foncière effectuent leur travail en 144 jours, contre 35 en 2010. Il y a matière à progresser, à moderniser et à sécuriser.

d'autoriser le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance pour la réforme de la publicité foncière, qui, je le rappelle, constitue un enjeu

Comme vous le savez certainement tous dans cet hémicycle, l'Alsace-Moselle a un droit local de la publicité foncière. cet article que nous examinons renvoie à une ordonnance la réforme du droit de la publicité foncière au niveau national, je me permets de demander au Gouvernement de tenir compte des spécificités de l'Alsace-Moselle en la matière. Je suis sûr que je serai entendu ! La parole

de l'étendue des sujets abordés dans le présent projet de loi, on s'étonne peu de retrouver ici un dispositif traitant de la mutualisation des fonctions support d'établissements publics de l'État. L'objectif affiché peut paraître de prime abord positif : mutualiser les moyens nécessaires à l'exercice commun d'activités. Mais notre inquiétude porte sur le fait que cette proposition n'est qu'un nouveau moyen de faire des économies d'échelle, sous couvert de simplification, et donc de réduire les moyens consacrés aux établissements publics de l'État qui réaliseraient de telles mutualisations.

429. En complément de ce que vient de dire notre collègue Michelle Gréaume, il est évident que, s'agissant de cet article 66, le Gouvernement n'a pas mis à profit la période qui a suivi la censure du Conseil constitutionnel pour préciser ses intentions,

des fonctions support des établissements publics. Je rappelle que les établissements publics ont cette particularité d'être territorialisés géographiquement et de ne pouvoir agir en dehors de leur ressort.

Ainsi, dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, il peut être utile de préciser un tel critère d'accessibilité pour pouvoir imposer ensuite plus facilement aux autorités administratives sa prise en compte.

», cet article ouvre la voie à la réalisation financière du patrimoine immobilier de la Monnaie de Paris. Je pense notamment à l'établissement de Pessac, qui était valorisé à 12,6 millions d'euros dans le rapport financier pour 2020.

l'érosion de l'usage des espèces dans les transactions. Mais on sait que cette dématérialisation

pour l'avenir de la Monnaie de Paris, en valorisant ses collections historiques et en trouvant de nouvelles missions. La voie choisie ne nous paraît pas opportune : c'est pourquoi nous proposons la suppression de l'article.

Je tiens à vous dire, monsieur le sénateur, que ce projet a reçu le soutien du corps social de cette entreprise qui a un caractère, comme on le sait, un peu particulier, les représentants des salariés présents au conseil d'administration. Un vote unanime en faveur

qui met en place, au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le comité social d'administration, en lieu et place des trois instances de concertation actuelles prévues à l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, à savoir- je le rappelle, mais vous les connaissez tous -le comité technique, le comité social et économique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. reprend à ce titre les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Notre groupe s'oppose à cette « simplification » et à la transformation des comités, qui sont des espaces de dialogue social importants pour les agents de la fonction publique.

sans consultation préalable des divers syndicats, il semble problématique de demander au législateur de voter une telle mesure. Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Quel est

J'estime que c'est une voie plus efficace de dialogue social, comme on peut l'avoir aujourd'hui dans les entreprises ou dans d'autres structures de l'État.

Il me semble difficile de trouver pour quelles raisons l'ANCT, qui, au même titre que tous les établissements publics, est bien couverte par cette disposition, en serait exemptée et en quoi elle serait différente des autres établissements et agences où cette même logique de réforme s'applique.

les personnels de l'ANCT ont eu connaissance, lors d'une réunion du comité technique et du comité social et économique, organisée à la fin de l'année 2020, de ces dispositions. Pour l'ensemble de ces raisons, et dans une logique d'harmonisation et d'équité entre les différents établissements publics de l'État, nous sommes attachés, avec Jacqueline Gourault

bis Mesdames les ministres, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin de poursuivre l'examen de ce texte jusqu'au vote sur l'article 73 .

Ce chapitre VII, entièrement dédié à la transparence et à l'agilité des entreprises publiques locales, était très attendu par de nombreux élus locaux engagés dans ce mode de gestion. Constitué de onze articles, dont sept nouveaux émanant de nos rapporteurs, il améliore leur fonctionnement, sans

Les articles traitent donc de contrôle de gestion, de transparence, de déclaration d'intérêts, de fiscalité, de déontologie, de la rémunération des dirigeants, de statut des membres élus, etc.

ou enfin à finaliser la gamme des entreprises publiques locales en Nouvelle-Calédonie. Hélas, trois fois hélas, cinq de ces amendements, largement cosignés par mes collègues, ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution, pour certains parce qu'ils incitaient à la dépense. Aussi, nous n'en discuterons pas ce soir, alors que nous espérions pouvoir être suivis par nos collègues, mais aussi par le Gouvernement, sur ces propositions d'évolution et de modernisation de l'action publique locale. Notre objectif était pourtant de tendre vers cet ajustement législatif et réglementaire qui permettrait à ces entreprises d'agir sur des problèmes d'éthique spécialisés, de continuer de travailler sereinement avec les pouvoirs publics et de s'adapter aux phases de décentralisation que nous connaissons ou appelons de nos voeux, dans l'intérêt des territoires et de leurs habitants. L'amendement

transparence et sécurité, sans oublier qu'il s'agit d'économie, même si c'est de l'économie mixte, qui concerne essentiellement les collectivités. Il y a donc des temps d'action, des temps de réactivité, des délais à respecter.

diminué le contrôle des assemblées délibérantes. Nous avons essayé d'être exigeants, mais réalistes et pragmatiques. Demander l'avis de toutes les collectivités membres d'une EPL avant de prendre une décision

délibérante. Nous proposons de compléter l'article pour couvrir les spécificités des sociétés publiques locales auxquelles s'applique cette partie du code en prévoyant que ce rapport pourra, le cas échéant, dresser un état des dispositifs mis en oeuvre par toute collectivité ou groupement actionnaire pour exercer son contrôle analogue. Compte tenu du niveau de précision de l'article 70 ainsi complété, il apparaît superfétatoire de préciser son contenu par décret, l'objectif de renforcement de la transparence autour de ce rapport étant déjà largement atteint.

pour préciser le contenu du rapport des mandataires des collectivités territoriales. Vous l'avez dit, la Fédération des EPL a élaboré un Livre blanc très

Comme je le disais précédemment, la rédaction initiale du Gouvernement tenait compte des recommandations de la Cour des comptes en renforçant le contrôle des collectivités locales sur les prises de participation (SEM) dans d'autres sociétés. Elle intégrait notamment une sanction de nullité en cas de défaut d'accord de la collectivité. La commission des lois a

au regard des risques financiers qu'elles impliquent. Il s'agit de protéger les collectivités. La filialisation ne doit pas conduire les EPL à s'écarter de leur mission. Pour les participations indirectes dans les sociétés commerciales comme civiles, le Gouvernement propose de conserver le seuil de 10 % adopté par la commission. Cependant, dans ce cas, il faut que l'ensemble des collectivités actionnaires soient consultées. C'est le sens de la rédaction proposée.

qui permet d'apporter de la souplesse et de la sécurité.

actionnaires d'une SEM a le pouvoir de s'opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d'une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l'organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaires se prononce sur cette opération. Compte tenu des modalités de fonctionnement internes des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce contrôle subordonne ces prises de participation à des contraintes de délai qu'il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Or l'article 70 du projet de loi, dans la rédaction rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit d'étendre cette contrainte procédurale à toute prise de participation indirecte, quel que soit le lien existant entre la SEM et la société qui prend la participation. Un tel formalisme est tout à fait injustifié, s'agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles des personnes publiques ne participent pas. D'un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l'accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d'autres sociétés ou de groupements d'intérêt économique (GIE), compte tenu, d'une part, de la difficulté qu'il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l'accord est requis, et, d'autre part, du délai nécessaire pour obtenir l'ensemble des délibérations afférentes. D'un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s'opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d'entreprendre, qui a valeur constitutionnelle. Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public. C'est la raison pour laquelle, au travers de l'amendement n° 1546 rectifié , nous souhaitons des prises de participation indirectes à celles qui conduisent la SEM à prendre le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société faisant l'objet de la prise de participation. Pour ce qui concerne l'amendement il convient de se référer à l'article L. 233-2 du code de commerce, qui définit la notion de prise de participation : lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction de capital comprise entre 10 % et 50 %, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde. Tel qu'il est rédigé, le dispositif de contrôle prévu à l'article 70 s'appliquerait dans tous les cas où la prise de participation, directe ou indirecte, conduit à la détention d'au moins 10 % du capital de la société qui en a fait l'objet. En conséquence, toujours dans le même souci de ne pas soumettre des prises de participation indirectes

Cet amendement vise à imposer la nomination d'un commissaire aux comptes dans toutes les filiales et les groupements d'intérêt économique, en instaurant, comme pour les autres entreprises, un dispositif applicable uniquement aux filiales significatives de sociétés d'économie mixte locales et aux GIE dépassant les seuils de la loi Pacte. Au regard de l'enjeu, l'obligation pour les filiales de petite taille de se doter d'un commissaire aux comptes en propre n'apparaît pas nécessaire, d'autant plus que les commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte mères ont déjà la possibilité de consulter les comptes de ces filiales. Les sociétés d'économie mixte en rendent compte dans leur rapport de gestion communiqué aux organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires. L'augmentation sensible des charges de de gestion que représenterait le fait de se doter d'un commissaire aux comptes pour les petites filiales serait de l'ordre de 3500 euros à 5 000 euros. Cette obligation apparaît en outre disproportionnée, d'autant que ces filiales sont souvent constituées pour des projets ponctuels, comme des opérations de réhabilitation d'ensembles immobiliers destinés à être loués à loyer modéré.

l'article 71, pour les commissaires aux comptes d'une SEM de signaler aux collectivités territoriales et à leurs groupements actionnaires, à la chambre régionale des comptes et aux représentants de l'État dans le département, les irrégularités ou inexactitudes qu'ils auraient détectées dans les comptes de cette SEM. Ce dispositif de signalement n'apparaît pas nécessaire au regard du cadre déjà prévu par le code de commerce pour les contrôles effectués par les commissaires aux comptes. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes doivent déjà signaler, lors de l'assemblée générale ou de la réunion de l'organe compétent la plus proche, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. S'agissant des interventions auprès d'une entité d'intérêt public, ils sont invités à enquêter, conformément au dispositif de l'article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont déjà l'obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. Enfin, aux termes de l'article L. 234-1 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d'une société d'économie mixte relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit en informer le président du conseil d'administration ou du directoire. À défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter par un écrit, dont une copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou du directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.

que les recommandations de la Cour des comptes pointaient le nécessaire renforcement du rôle du commissaire aux comptes, ce à quoi nous avons procédé. Nous avons trouvé un point d'équilibre entre le texte du Gouvernement

La commission des lois a souhaité supprimer la sanction de nullité des actes non transmis par les EPL, en lui substituant une possibilité pour le préfet de demander par voie de justice aux dirigeants d'une EPL de lui communiquer lesdits actes. Cette mesure paraît tout d'abord difficilement applicable, dans la mesure où, en cas de non-transmission d'un acte au préfet, celui-ci n'a précisément pas les moyens de savoir que l'obligation n'est pas respectée. Il est fortement souhaitable que cette obligation de transmission, d'ores et déjà requise par la loi, soit respectée. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de la Cour des comptes. Il revient à l'EPL qui se soustrait à ses obligations d'en supporter la responsabilité. L'amendement vise donc à rétablir la sanction de nullité initialement prévue en cas de non-transmission des actes. Le régime de la nullité, en droit des sociétés, est plus adapté à la nature des EPL qu'une mesure privant d'effet un acte non transmis, à l'instar de ce que prévoit le contrôle de légalité.

engagées. Au final, la situation serait extrêmement difficile pour les acteurs économiques. Il nous a semblé préférable de choisir une autre sanction, qui est la mise en demeure par le préfet de transmettre les actes que l'EPL aurait dû transmettre,